sujet est particulièrement sensible. Au total, dans le projet de loi de finances pour 2023, les transferts financiers de l'État au profit des collectivités territoriales s'élèveraient à 107,6 milliards d'euros, répartis comme suit : 53,1 milliards d'euros pour les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, 39,3 milliards d'euros pour la fiscalité transférée et 14,4 milliards

l'inflation comprime actuellement la dépense publique en diminuant la valeur des concours financiers de l'État aux collectivités. La loi de programmation des finances publiques a arrêté une trajectoire de réduction des concours financiers de l'État en volume. un rationnement qui ne dit pas son nom ! Certes, les dotations et le FCTVA augmenteront bien de 2,6 % en euros courants. Mais, en tenant compte de l'inflation, c'est une ponction de 4,1 milliards d'euros de 2023 à 2027 que vous avez inscrite dans la loi.

à chaque budget ! Il est donc impératif d'indexer dès à présent la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales sur l'inflation

évoluer au même rythme que l'inflation. Deux chiffres témoignent de l'importance d'une telle mesure. Entre 2017 et 2021, la non-indexation a représenté un manque à gagner de l'ordre

Ensuite, les dotations ne sont pas des subventions de l'État. Elles sont non pas un don, mais un dû ! C'est la contrepartie, à l'euro constant près, soit de la nationalisation d'une fiscalité jusqu'alors locale, soit d'un transfert de charges de l'État vers les collectivités. Notre principe constitutionnel de libre administration des collectivités ne doit plus être bafoué. Ne pas garantir en euros constants les recettes censées appartenir aux collectivités, le produit du résidu de fiscalité locale et, surtout, des dotations qui s'y sont substituées, remet en cause pour chacune d'entre elles- mes collègues l'ont déjà souligné -un équilibre déjà précaire. De plus,

aux préoccupations légitimes des maires et des présidents d'intercommunalités, pour qui le coût des dépenses contraintes a augmenté de manière exponentielle. En effet, à l'instar de la population, les communes subissent de plein fouet l'inflation

Par vos réformes, vous siphonnez de manière systémique leurs recettes, plaçant ainsi les communes sous perfusion de dotations, que vous pouvez moduler de façon discrétionnaire. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'être à la hauteur des besoins, ce qui suppose d'émettre un avis favorable sur notre amendement.

retire, monsieur le président.

Monsieur le ministre, je peine à comprendre si vous saisissiez bien les enjeux qui se présentent à nos collectivités territoriales aujourd'hui.

et qui pourraient représenter encore davantage ? Nous proposons également de supprimer les minorations des dotations de l'État aux collectivités, avec la baisse prévue de 45 millions d'euros en rognant sur les compensations des départements et des régions. Les trois amendements

En 2022, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et la dotation pour transferts de compensation d'exonération de fiscalité directe locale (DTCE) des régions se montent respectivement à 467 millions d'euros et à 15,8 millions d'euros et constituent des ressources à part entière de leur budget. Entre 2017 et 2022, la DCRTP et la DTCE des régions ont respectivement enregistré une baisse de 207 millions d'euros et de 108 millions d'euros

totale d'impôt sur les bénéfices, sur le revenu, sur les cotisations sociales et d'impôts locaux, ainsi que d'une exonération dégressive les trois années suivantes. Afin d'éviter les effets d'aubaine et les stratégies d'optimisation fiscale, il a également été mis en place plusieurs dispositifs anti-abus. anti-abus. Une application stricte de ces clauses anti-abus pourrait paraître suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins désirant s'installer durablement dans une ZRR. Or il n'en est rien, puisque l'on observe sur les territoires des phénomènes « d'installations et de désinstallations » périodiques durant les huit années d'exonération. C'est ce que

même partiellement, sa patientèle, ne peut pas être analysée comme une création, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du bénéfice de l'exonération. Il est donc proposé par cet amendement d'ajouter à l'exonération un ultime dispositif anti-abus en ne permettant la la réinstallation d'un médecin déjà installé dans une ZRR qu'à la condition d'être à plus de 50 kilomètres de son ancien cabinet. Quel est l'avis de Sur le fond, l'objectif de limitation des abus est évidemment souhaitable. Toutefois, le droit existant et la doctrine administrative permettent d'éviter que des entreprises ne délocalisent leurs activités

L'objectif des ZRR, lors de leur création, était bien de favoriser l'installation de toute activité économique dans les territoires souffrant d'un manque d'attractivité. Madame la sénatrice, je suis d'accord avec vous, il apparaît- cela a été documenté par un certain nombre d'études et de rapports -que les aides fiscales de ce zonage conduisent parfois à des effets d'aubaine, notamment pour certaines professions qui relocaliseraient plus facilement leur activité pour bénéficier des exonérations.

Malgré les politiques actuelles menées en faveur de la revitalisation des campagnes, de nombreuses communes rurales éprouvent les plus grandes difficultés à préserver les dernières activités économiques encore présentes. Il apparaît nécessaire, voire impérieux de stimuler le tissu de petites entreprises qui se trouvent sur ces territoires en les incitant à s'y maintenir et de soutenir pleinement la viabilité économique des activités de nos campagnes, qui, si elles demeurent majoritairement modestes, apportent des services essentiels dans les territoires ruraux. telle mesure répondrait à deux enjeux : d'une part, à l'enjeu économique, en permettant aux activités concernées de se maintenir ou en aidant les employeurs à recruter et à afficher des offres plus attrayantes, soutenant l'emploi dans ces zones fragiles ; d'autre part, à l'enjeu écologique, en proposant des emplois et des services au plus proche des bassins de vie ruraux en diminuant les temps de trajet, les émissions polluantes, mais aussi les frais inhérents aux déplacements. Dans cette perspective, la mesure d'exonération proposée contribuera, dans les communes volontaires, à baisser les charges fiscales locales des entreprises fragilisées et à renforcer le développement économique dans les territoires ruraux.

secours (Sdis) ont besoin d'un financement croissant pour faire face à l'augmentation des interventions liée à différents facteurs, comme la pénurie de médecins et le réchauffement climatique, qui ne vont que s'aggraver avec le temps, il paraît nécessaire que la totalité de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) affectée aux départements pour les Sdis revienne réellement à ces derniers. L'accroissement des ressources des Sdis leur permettrait également d'améliorer leur équipement pour alléger les contraintes parfois excessives qui pèsent sur les communes en matière de défense extérieure

du 5 de l'article 1001 du code général des impôts, affectée à l'ensemble des départements et destinée à contribuer au financement des services d'incendie et de secours. Certes, le produit de la taxe a évolué. Pourtant, cette part n'a pas été corrigée depuis 2007 et reste néanmoins mécaniquement plafonnée, alors même que les services d'incendie et de secours font face, chaque année, à une augmentation continue de leur sollicitation opérationnelle pour garantir la protection et la sauvegarde de nos concitoyens, de nos entreprises et de l'environnement. Ainsi, à la lumière de l'année 2022, la question du financement des Sdis est aujourd'hui un sujet majeur de préoccupation, notamment pour les collectivités locales. Elle l'est aussi pour le nécessaire renforcement capacitaire des moyens matériels et humains de ces services, afin de leur permettre de prévenir et de lutter contre la multiplication et l'intensification des événements climatiques extrêmes liés au dérèglement climatique sur l'ensemble du territoire national. Une telle mesure constitue une première réponse immédiate au renforcement organisationnel et opérationnel de notre modèle de sécurité civile souhaité par le Gouvernement à la suite des événements climatiques extrêmes de l'année 2022. La

la « valeur du sauvé ». Cette vision consiste à prendre en considération tout ce qui a été sauvé par les sapeurs-pompiers- habitations, biens, forêts -et qui, par conséquent, ne fera pas l'objet d'indemnisation de la part des assurances. En un mot, les pompiers font économiser de l'argent aux assurances, et pas qu'un peu ! La dernière étude à notre connaissance réalisée par le Sdis des Bouches-du-Rhône évalue ce gain à 1,8 milliard d'euros pour l'année 2020. C'est probablement beaucoup plus pour cette année. Il semble dès lors logique que les assurances financent davantage notre modèle de protection civile. C'est un amendement de bon sens, défendu par de nombreux groupes

Mais il ne me semble pas forcément souhaitable de passer à côté des départements, qui sont les principaux financeurs des Sdis.

158 millions d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement et 38,5 millions d'euros sont prévus sur le programme « Sécurité civile » pour permettre de financer les pactes capacitaires entre l'État, les collectivités et les Sdis.

C'est une partie des ressources de ces services, qui s'élèvent à plus de 5 milliards d'euros. Les amendements présentés visent soit à transférer l'intégralité de la TSCA aux Sdis sans passer par les départements, soit de doubler la fraction de TSCA

à supprimer le critère de potentiel financier de la commune, ce qui ferait que toutes les communes de moins de 1 000 habitants pourraient en bénéficier. J'y suis défavorable, pour des raisons d'encadrement des finances publiques. On peut être une très petite commune,

à laquelle se trouvent confrontées les communes pour s'assurer contre le risque inondation. La piste d'un recours au fonds Barnier avait notamment été avancée. Le présent amendement a pour objet de proposer une solution dans le respect des règles de recevabilité de l'article 40 de la Constitution, qui s'opposent à ce qu'un abondement du fonds Barnier soit proposé par un amendement parlementaire. Cette solution consiste à instituer par prélèvement sur les recettes de l'État une dotation d'aide à l'assurance contre les inondations dans les territoires « dans lesquels il existe un risque d'inondation important ayant des conséquences de portée nationale ». La dotation servirait à rembourser au groupement de communes chargé de la compétence « défense contre les inondations » une part de la prime d'assurance. La perte de recettes pour l'État serait compensée dans une large mesure par un prélèvement sur les primes d'assurance contre les inondations. Il s'agirait donc, dans la même logique que le fonds Barnier, de faire jouer la solidarité nationale. Quel

en lieu et place de l'actuelle dotation budgétaire du même nom. La dotation budgétaire destinée à compenser les investissements en faveur de la biodiversité réalisés par les communes situées dans un parc naturel marin ou un site Natura 2000 a été instituée en 2019. Elle a été élargie aux communes situées dans un parc national en 2020 et aux communes situées dans un parc naturel régional en 2022. Son montant total a atteint 24,32 millions d'euros en 2022. Il est proposé de mettre en cohérence un dispositif modernisé de soutien aux communes sous la forme d'une dotation dont les crédits seraient répartis par le comité des finances locales selon les deux axes suivants. Il s'agit, en premier lieu, d'étendre le versement aux communes concernées par une zone de « protection forte lieu, pour les zones n'étant pas reconnues au titre du décret « protection forte », de reconnaître l'engagement des communes en faisant bénéficier de la dotation celles qui sont chargées de l'animation des démarches territoriales ou qui adhèrent à une charte d'espace protégé.

du FCTVA subsistent : l'année même de l'investissement, pour les communautés ; en année pour les collectivités ayant opté en 2019 pour ce régime ; en année pour les autres collectivités Il n'y a plus de raison que subsiste un régime en année . Il est donc proposé de supprimer ce régime au bénéfice du. Sur la période des cinq années, l'incidence globale est neutre, les dépenses en 2023 étant compensées par une baisse de dépenses étalées sur les quatre années suivantes. Quel

ses dépenses qui avaient toujours été prises en compte ne le sont désormais plus. À l'époque de la réforme, qui a produit des effets très positifs par ailleurs, il avait été décidé qu'elle serait à coût constant pour l'État.

un artifice vient perturber le dispositif : le potentiel financier est lié de manière artificielle à l'intégration fictive d'une partie des ressources de l'EPCI. Avec ce mode de calcul, on exclut du bénéfice

En 2022, ce coût a été estimé à 1,13 milliard d'euros. Le mécanisme d'aide adopté dans le cadre de la loi de finances rectificatives pour 2022 est beaucoup trop restreint et ne permet pas de compenser cette augmentation. Le coût du dispositif gouvernemental devrait s'élever à seulement 430 millions d'euros, et comprend également une compensation minime de certaines conséquences de l'inflation et des critères très restrictifs. environ 22 000 communes seraient potentiellement éligibles ; mais, selon l'AMF, les bénéficiaires devraient être moins nombreux. Une récente étude de la Banque postale indique que seulement 8 000 communes seraient en réalité concernées. La revalorisation du point d'indice, décidée par le Gouvernement, est financée par les collectivités employeurs, déjà largement mises à contribution. Elle va fortement peser sur les finances locales, qui finissent difficilement l'année 2022 l'épargne brute des collectivités serait en repli de 4,4 % cette année en raison de l'inflation, avec des dépenses de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes. Pour 2023, le coût de la revalorisation est estimé à 2,27 milliards d'euros. Les collectivités sont évidemment favorables à la revalorisation du traitement des agents publics, surtout au regard de la perte d'attractivité de ces emplois.

leurs conditions de travail et de rémunération difficiles et à un cadre d'emploi éclaté. Parfois, ce sont jusqu'à quatre mairies qui se partagent une secrétaire de mairie, avec tous les trajets que cela implique inévitablement. Quel est l'avis de la commission

supplémentaire très lourde pour les budgets des départements. Cette décision de revalorisation a été actée de manière unilatérale par l'État et a été imposée aux élus locaux et aux départements, finances sont déjà sous pression. Il n'est donc pas normal que ces derniers aient à supporter seuls le coût de la décision. Cette mesure de justice sociale fait suite à une première revalorisation de 1,8 % au mois d'avril dernier. Or l'impact économique de la nouvelle revalorisation de 4 % serait de 400 millions d'euros en 2022 et 800 millions d'euros en année pleine. Le coût pour les finances des départements serait donc de 120 millions d'euros pour 2022 et de 240 millions d'euros pour 2023 au titre du RSA. Il est essentiel de le rappeler, le RSA fait partie des compétences décentralisées que l'État s'est engagé à compenser. Or force est de constater qu'il ne le fait pas. En effet, sur les 11 milliards

Il est important de mettre en avant ces chiffres, car, concrètement, faire assumer aux départements la dépense sociale supplémentaire, c'est venir limiter encore un peu plus leurs marges de manoeuvre alors qu'ils sont pourtant des acteurs-clefs de la cohésion sociale. Une juste compensation de l'État s'impose. En conséquence, cet amendement prévoit de prolonger la compensation opérée sur les recettes de l'État au profit des départements qui a été adoptée au mois d'août 2022. Il tend ainsi à créer un nouveau prélèvement permettant d'assurer une telle compensation

La dotation de continuité territoriale (DCT) est un concours individualisé de l'État versé à la collectivité de Corse pour lui permettre de mettre en oeuvre le principe de continuité territoriale, tel qu'il a été défini en 1976, en organisant et finançant les dessertes maritime et aérienne liant la Corse au continent. Les modalités de versement de ladite dotation sont précisées à l'article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales. Depuis 2009, la dotation est gelée et n'évolue plus, restant établie à près de 187 millions d'euros. L'évolution des prix et l'envolée du coût du carburant et de l'inflation compliquent la tâche des compagnies délégataires, qui ne peuvent pas faire face au flux constant au flux constant de ces modulations sans que les montants de compensation évoluent dans les mêmes proportions. La DCT ne pouvant être majorée pour une question de recevabilité financière, il est proposé, à l'instar de ce qui a été établi lors du PLFR pour

au maître d'ouvrage délégué. De manière très concrète, des communautés de communes portant des opérations pour le compte des communes pouvaient percevoir le FCTVA. À la fin, le solde de l'autofinancement revenant

Ainsi serait promue l'économie de l'usage, de la fonctionnalité, généralement plus vertueuse en matière environnementale et économe en ressources.

nous, il convient de couvrir aussi les dépenses de fonctionnement, qui représentent une part importante de leur budget. La limitation aux seules dépenses d'investissement ne fait plus sens dès lors que certaines dépenses de fonctionnement des collectivités sont aussi incluses dans l'assiette Cette mesure, qui vise à plus de sécurité financière et d'équité, est demandée par certains Sdis, à l'instar de celui de la Métropole de Lyon, que l'on appelle SDMIS. J'ajoute pour mes collègues de la majorité sénatoriale qu'un amendement similaire avait été déposé par les députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, mais qu'il n'a pas pu être examiné à cause

représenterait un coût majeur, 6 milliards d'euros, pour un effet limité. L'avancement du versement du FCTVA a été testé par l'État au moment de la crise de 2008 à 2010 comme une réponse pour encourager l'investissement local.

L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les collectivités territoriales ne peuvent pas bénéficier des attributions du FCTVA pour leurs dépenses d'investissement en matière de bâtiments mis à disposition de l'État pour les besoins de la gendarmerie, à moins que ceux-ci ne soient mis à disposition de l'État à titre gratuit. Compte tenu des montants de ce type d'opérations, qui ont un poids considérable pour le budget des communes, notamment en ce moment, l'absence de récupération de la TVA n'est pas une option envisageable. En effet, les loyers couvrent déjà rarement la totalité de la charge de l'emprunt, et, comme ils sont fixes, ils ne permettent pas d'anticiper l'entretien des bâtiments, qui reste de ce fait à la charge de la commune. suite de la récente réforme de l'automatisation de la TVA, il semblerait que la récupération soit désormais possible pour les communes, à condition que celle-ci ne soit pas récupérable par voie fiscale. Un doute subsiste cependant sur l'éligibilité des dépenses, puisque les collectivités territoriales peuvent récupérer la TVA par la voie fiscale en appliquant celle-ci, sur option, aux loyers de la caserne. De plus, en tout état de cause, l'article L. 1615-7 du CGCT indique toujours que la récupération n'est possible que si le bâtiment est mis à disposition à titre gratuit. Cet amendement a donc pour objet de graver dans le marbre qu'il est permis aux communes de récupérer la TVA. Cela assurerait un allégement du coût restant à leur charge, et ce quel que soit le mode de location ou de mise à disposition

tiers. S'il y a un loyer qui est assujetti à la TVA, cela n'entre pas dans le FCTVA, mais la collectivité bénéficie d'une récupération par voie fiscale.

leur entretien, ce qui représente pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leurs capacités financières. Lorsque les conséquences sont aberrantes, il est urgent de corriger ou d'adapter notre droit, surtout dans un domaine touchant aussi étroitement à la sécurité des personnes et des biens que la biens que la lutte contre l'incendie. Cet amendement vise à instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75 % des dépenses d'équipement en points d'eau contre l'incendie et des dépenses consacrées à leur entretien. Seraient également couvertes, car se rapportant à des opérations qu'il convient évidemment d'accompagner, les dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie. Quel La lutte contre les incendies est une compétence des communes et des départements. Pour ma part, je pense qu'il ne revient pas à l'État de financer les dépenses réalisées à ce titre.

? Avis défavorable, pour plusieurs raisons. D'abord, il existe actuellement des dispositifs de soutien à l'investissement local

16 millions d'euros ont été attribués au titre de la DETR pour le financement de 1 029 opérations liées à la défense contre les incendies, et plus de 3 millions d'euros ont été attribués au titre de la DSIL pour 43 opérations dans ce même domaine. J'ajoute que les dépenses de ce type sont éligibles au FCTVA.

par propriétaire. Des centaines de propriétaires peuvent se manifester, et des centaines de communes rurales sont concernées. Certes, l'article L. 2225-2 du CGCT dispose que les communes sont « chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie », mais c'est impossible à financer et très compliqué techniquement à mettre en oeuvre. D'où cette solution

Cependant, depuis de nombreuses années, les élus insulaires demandent une réforme de cette affectation. En effet, elle ne correspond à aucune logique économique, selon les mots mêmes, d'ailleurs, de l'administration fiscale française, puisqu'elle subordonne l'équilibre du budget de la CDC à l'évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique, ainsi qu'à l'évolution des comportements au sein de la population corse. Aussi, le présent amendement de bon sens vise à transférer, selon les recommandations que vous n'êtes pas censés ignorer, censés ignorer, les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale, et, condition, à remplacer cette recette par une fraction de produit de la TVA, de façon similaire à la dotation globale de décentralisation.

des ressources (FNGIR) vise à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes. Toutefois, d'année en année, la déconnexion entre les raisons de sa création et la réalité du tissu économique est de plus en plus importante. En outre, la réduction des leviers fiscaux dont disposent les collectivités accroît fortement son impact dans leur budget. La fixité du FNGIR est source d'importantes inégalités. Le Gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à réformer le FNGIR et à mettre ainsi fin à cette injustice. L'article 79 de la loi de finances pour 2021 avait apporté une première réponse provisoire en mettant en place un prélèvement sur les recettes de l'État à destination des communes contributrices

Toutefois, cette double conditionnalité se traduit par un petit nombre de communes réellement concernées et désavantage les petites communes dont la perte de base de CFE peut être inférieure à 70 %, mais pour lesquelles le prélèvement FNGIR représente parfois plus de 10 % des recettes réelles de fonctionnement, ce qui grève fortement leur budget. Aussi, cet amendement vise à réduire l'effet de seuil défavorable aux petites communes par une extension du dispositif mis en place dans la loi de finances pour 2021, en abaissant la condition de perte de base de CFE à 50 % pour les communes dont le prélèvement FNGIR représente au moins 10 % des recettes réelles de fonctionnement. cet amendement vise à réduire l'inégalité que j'évoquais pour les quelques dizaines d'EPCI concernés, en compensant partiellement leur contribution au FNGIR par un plafonnement à hauteur de 100 % de leurs recettes de fiscalité économique.

en 2021, la restauration collective concernait 10 millions de personnes chaque jour. Ce sont 3,1 milliards de repas qui sont servis chaque année, pour un chiffre d'affaires global de 18 milliards d'euros. La restauration collective offre ainsi un débouché très important pour nos filières agricoles, les collectivités territoriales subissent de plein fouet les crises successives et l'inflation. Ainsi, le coût moyen d'un repas se situait avant ces crises aux alentours de 2 euros.

le principal, voire le seul repas équilibré de la journée. D'autre part, l'inflation risque de mettre un coup d'arrêt aux efforts des collectivités en matière d'achat de produits locaux et durables, ce qui pénalise la transition agroécologique et prive les agriculteurs de débouchés. à tous, dite loi Égalim, avait fixé à la restauration collective des objectifs d'approvisionnements de qualité, locaux et bio. Or ceux-ci ne sont malheureusement pas atteints

Entre les différentes lois, il existe parfois un interstice où elles interviennent en concurrence. Nous en avons là un cas d'espèce. Ainsi, le maire de la ville de Grigny, M. Philippe Rio, avait interpellé le Président de la République dès 2019 sur une sur une situation profondément injuste touchant, d'après une étude réalisée par un cabinet, une petite quarantaine de communes de France, qui connaissent une augmentation démographique plus importante que la moyenne, tout en étant tributaires de ressources moins élevées qu'ailleurs. C'est le fameux « 30 % de capacités financières en moins pour 30 % de besoins en plus », identifié par le rapport Borloo du mois d'avril 2018 sur les quartiers prioritaires de la ville.

d'un ajustement du montant du droit à compensation aux régions résultant du transfert de la compétence d'autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres.

par les collectivités locales, dans la mesure où il définit le filet de sécurité énergie dans sa version 2023. Ce filet vient compléter le dispositif de bouclier énergétique qui protège les particuliers et les collectivités les plus petites avec les tarifs réglementés de vente. Je pense qu'il est utile de vous transmettre les interrogations de beaucoup d'élus locaux, qui se demandent pourquoi ces tarifs réglementés ne peuvent pas profiter à plus de collectivités locales

dont deux tiers peuvent être éligibles au tarif réglementé et elles ne représentent que 15 % de la consommation électrique.

À bien des égards, le dispositif est même plus restrictif, en ne compensant que les dépenses d'approvisionnement en énergie, et non plus les dépenses d'achat de produits alimentaires ou la revalorisation du point d'indice

une compensation instituer un bouclier énergétique au profit des communes, de leurs groupements, des départements et des régions. Il est proposé que l'État compense à hauteur de 50 l'augmentation des dépenses énergétiques subie par les communes, leurs groupements, les départements et les régions lorsque celle-ci est, en 2023, supérieure à la moyenne lissée des dépenses énergétiques engagées en 2017, 2018 et 2019. L'année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence compte tenu de l'incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur les dépenses en énergie des collectivités territoriales.

des recettes de fonctionnement pour déclencher une prise en charge, une fois ce seuil dépassé, à hauteur de 50 % du dépassement. Nous proposons d'abaisser ce seuil de déclenchement à 40 %.

est envisagé de bien tenir compte des dépenses et recettes, mais en retirant le critère de dégradation de la situation financière de la commune dans le cours de l'année.

Enfin, les auteurs de certains amendements font la comparaison sur la situation financière et la perte d'épargne brute non pas entre 2022 et 2023, mais entre 2021 et 2023. Je pense que c'est intéressant,

est à M. Fabien Genet. Je suis assez sensible au discours de vérité que vient de tenir le ministre, car j'ai le sentiment qu'on ne l'entend pas dans beaucoup de bouches ministérielles ces derniers temps.

la fin de l'année 2023 sera très compliquée. Ce sous-amendement vise ainsi à prendre en considération le différentiel entre 2021 et 2023, et non pas entre 2022 et 2023. En effet, pour les collectivités qui auront franchi une première marche

aider. Autrement dit, avec votre système, si une collectivité franchit une marche importante en 2022, elle pourrait être aidée par le filet de sécurité 2022, mais ne plus rien toucher en 2023, alors même

des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain enregistrée en 2023 devrait être calculée en comparaison de l'année 2021, et non de

L'acompte serait alors versé non plus avant le 30 septembre, mais dans les deux mois suivant la demande de la collectivité ou du groupement.

: La parole est à Mme Sylviane Noël. Lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a intégré au titre de l'année 2023 un dispositif visant à soutenir les collectivités territoriales confrontées à une situation de forte inflation de leurs dépenses d'énergie. En l'état, ce dispositif profiterait aux collectivités qui qui auront subi en 2023 une perte d'épargne brute supérieure ou égale à 25 % et dont la hausse des dépenses d'énergie sera supérieure à 60 % de la progression des recettes réelles de fonctionnement. Le plafond de perte d'épargne brute supérieure ou égale à 25 % est trop élevé et n'englobera pas assez de communes, qui souffrent pourtant de ce contexte inflationniste. Il est donc proposé par cet amendement d'abaisser la perte d'épargne brute à 10 %, afin d'élargir le nombre de communes et de groupements bénéficiaires de la dotation. L'amendement n° I-1295,

2021, au lieu de l'année 2022. Il est également proposé de rehausser le seuil d'épargne brute retenu, afin de tenir compte de la baisse enregistrée en 2022 et en 2023.

consacrer quelques instants. Je remercie le rapporteur général de ses explications. Monsieur le ministre, nous essayons ici de faire

qui écrivait : « Mes crimes c'est avant de les commettre que j'aurais pu les regretter. » En l'espèce, il n'y a pas de crime, mais peut-être des erreurs qui pourraient se révéler funestes.